des difficultés d'insertion professionnelle ou des tensions existant sur le « marché du logement », le rattachement des enfants majeurs, mariés ou non, est l'une des réponses fiscales proposées par notre droit. La situation concerne environ 1,7 million de foyers fiscaux et le rattachement coûte 1,9 milliard d'euros au Trésor public, soit une incidence fiscale d'un peu plus de 1 000 euros par foyer fiscal concerné. On est donc assez loin de la niche fiscale génératrice d'un avantage indu ou exorbitant ... Cet amendement se détermine avec simplicité, en cohérence avec l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu que nous avons indiquée lors de la discussion de l'article. Il s'agit tout simplement de procéder au relèvement du seuil de plafonnement des effets du rattachement,

En proposant, comme nous le faisons, de modifier la progressivité des tranches du barème, nous poursuivons l'ensemble des objectifs ainsi définis. La mesure que nous préconisons est susceptible de dégager des marges de manoeuvre pour les finances publiques, tout en répartissant la charge fiscale au plus près des capacités contributives de chacun et chacune. Au-delà de l'examen de notre proposition, ce qui est en question, c'est bel et bien le fait que l'impôt sur le revenu, dans notre pays, est marqué par une forte concentration des revenus imposables, qui traduit la réalité des inégalités sociales, de patrimoine et autres, ces inégalités affectant également la situation générale du pays et son économie en particulier. Pour vérifier la réalité de ces inégalités, un simple examen des données officielles, présentes sur le site du ministère, suffit. Ainsi, en 2016, 749 000 foyers fiscaux ont déclaré un revenu supérieur à 100 000 euros annuels- ils cumulent plus de 140 milliards d'euros de revenus soumis au barème, soit une moyenne proche de 190 000 euros par foyer, tout de même -et acquitté 28 milliards d'euros d'impôt sur le revenu, soit environ 20 assez loin de l'impôt « confiscatoire ». À l'autre bout de la chaîne, si l'on peut dire, un peu plus de 14 millions de foyers fiscaux ont déclaré moins de 15 000 euros annuels, pour un revenu total de 107 millions d'euros environ, soit un revenu moyen de moins de 7 500 euros.

En l'espèce, il est prévu de rétablir la tranche de l'impôt sur le revenu à 5,5 %, supprimée en 2014, afin d'élargir l'assiette. En

par la loi de finances pour 2015 a été en partie responsable de cette évolution, qui fragilise le statut de l'impôt sur le revenu, lequel devrait rester l'impôt citoyen par excellence. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en son article XIII, dispose : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable, inférieur à 6 114 euros annuels, doivent continuer à ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu, il importe que ce dernier soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Au-delà de la mesure ponctuelle, il s'agit de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'État et les citoyens. Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2017.

l'effet incitatif de certaines dépenses fiscales destinées à soutenir des acteurs économiques ou des acteurs sociaux qui opèrent dans nos territoires. Je partage le sentiment du rapporteur général sur

le Président de la République et le Gouvernement étant assez ouverts à la discussion, y compris sur des sujets aussi anciens que celui-là.

de faire baisser la pression fiscale- c'est l'autre argument que j'emploierai pour demander le retrait de cet amendement -, mais également de construire un édifice fiscal qui soit plus incitatif et qui rémunère justement les prises de risques

J'entends l'argument qui consiste à dire que le consentement à l'impôt sera d'autant mieux établi que la base de la population qui y consentira et le paiera sera large. Toutefois, les foyers les plus modestes participent déjà

M. Éric Bocquet, pour explication de vote. Avec ces trois amendements, nous sommes déjà au coeur du débat, et c'est bien qu'il s'engage. Je voudrais vous dire à quel point nous ne sommes pas des extrémistes de l'impôt sur le revenu.

En outre, l'annonce de la mise en oeuvre de la retenue à la source va sans doute faire naître, entre les salariés d'une même entreprise, bien des interrogations, singulièrement du fait de l'application du fameux quotient familial. Pour des raisons diverses, le quotient familial d'un foyer fiscal peut connaître une majoration d'une demi-part : celle-ci est, par exemple, liée à la situation de santé du contribuable, au service qu'il a rendu à la Nation- c'est le cas des anciens combattants -ou encore au fait qu'il a assumé seul la charge de l'éducation d'un ou plusieurs enfants. La demi-part des personnes seules

liées au quotient familial, qui prend en compte les situations réelles des ménages, coûtent au total un peu plus de 2 milliards d'euros au budget de la Nation, pour plus de 5 millions de contribuables. Ce dispositif constitue donc un élément de la politique sociale de la Nation, mais, pas plus que la suppression de l'exonération des majorations de pension, les mesures prises pour réduire leurs coûts ne se sont traduites par un renforcement des moyens de ladite politique. Tel est le sens de cet amendement. L'amendement

qui propose une revalorisation sélective du quotient familial selon la situation des contribuables concernés, je dois dire que le présent projet de loi de finances permet une revalorisation identique au taux de l'inflation- plus 1 %-de tous les plafonds et de toutes les demi-parts, notamment celles pour les invalides, les anciens combattants et les veuves. Il me paraît plus juste de procéder de la sorte, de façon générale. Avec la proposition du Gouvernement, le plafond du quotient augmente déjà de 15 euros

Les économies dégagées ont permis de maintenir le niveau des prestations, notamment pour les allocations familiales. Votre proposition remettrait en cause, en partie, l'équation financière de ce choix.

Pour un couple marié avec deux enfants, le plafonnement s'applique uniquement à ceux dont le revenu déclaré est supérieur à 5 930 euros par mois pour l'imposition des revenus de l'année 2016. Vous l'aurez compris, il y aura d'autres voies et moyens- nous aurons l'occasion d'en débattre -pour améliorer le pouvoir d'achat

d'avoir des enfants et de contribuer ainsi à la vitalité de notre pays et ceux qui- heureusement, ils sont de moins en moins nombreux ; c'est d'ailleurs un état d'esprit qui s'efface -, choisissent de ne pas avoir d'enfant

La convention de 1961 portant sur les fonctionnaires internationaux a aujourd'hui plus de cinquante-six ans. Alors que nous venons de parler d'une répartition plus juste des richesses et d'une contribution de chacun au budget des nations,

et qu'il serait opportun de réfléchir, malgré tout, à une contribution des fonctionnaires internationaux au fonctionnement des États dans lesquels ils vivent.

En effet, conformément au 8° de l'article 81 du code général des impôts, les indemnités journalières, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit, sont exonérées de l'impôt sur le revenu. En revanche, les indemnités journalières et les rentes d'incapacité permanente servies par le régime d'accident du travail des exploitants agricoles sont passibles de cet impôt. Il apparaît que cette imposition, même compensée, entraîne de vraies difficultés pour les exploitants agricoles,

la sénatrice, vous le savez, le Gouvernement est évidemment sensible aux risques auxquels les agriculteurs sont exposés dans le cadre de l'exercice de leur travail.

d'hébergement en établissement de long séjour. En l'état actuel des choses, il existe deux dispositifs bien connus : la réduction d'impôt accordée au titre des emplois dits familiaux et la réduction d'impôt liée aux dépenses d'hébergement en établissement de long séjour. Le premier de ces dispositifs intéresse plus de 3,8 millions de ménages, ce qui n'est pas du tout négligeable, et devrait coûter 4,74 milliards d'euros en 2018, faisant de cette dépense fiscale l'une des plus importantes du budget. Nous devrions donc passer d'une réduction d'environ 636 euros par ménage et par an à un crédit d'impôt environ deux fois plus important. Le second représente une dépense fiscale de 288 millions d'euros, au bénéfice d'un peu plus de 460 000 ménages, soit une réduction d'impôt moyenne de 620 euros par ménage et par an. Par conséquent, nous avons, d'un côté, un dispositif plutôt encore sous-dimensionné au regard des besoins, avec une dépense annuelle moyenne de 3 000 euros environ pour un plafond de 10 000 euros, et, de l'autre, un dispositif, à l'inverse, plutôt surdimensionné, avec moins de 1 500 euros de dépenses retenues pour un plafond minimal de 12 000 euros. Les dépenses d'hébergement en établissement de long séjour s'élèvent à près de 8 milliards d'euros pour environ 400 000 ménages, soit une dépense moyenne de près de 16 700 euros par ménage, bien supérieure, donc, au plafond de 10 000 euros. Un certain nombre de familles modestes, confrontées au problème de l'accompagnement du vieillissement de leurs aînés, se trouvent aujourd'hui contraintes de recourir au placement de leurs parents sans pouvoir réellement bénéficier d'une prise en compte, même limitée, de leur situation. leur situation. Nous proposons donc de procéder à la transformation en crédit d'impôt de la réduction d'impôt relative aux dépenses d'hébergement en établissement de long séjour, eu égard au caractère très imparfait encore de la solidarité nationale en la matière.

mais je pense que vous auriez dû prendre en compte cet amendement,

la réponse en matière de prise en charge de la dépense n'est pas que fiscale. Voilà quelques jours, j'étais encore président d'un conseil départemental, et il y a ici des élus départementaux qui savent que les départements

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la généralisation de ce crédit d'impôt, étendu en janvier 2017 à tous les contribuables. Cet amendement, s'il est voté, permettra de baisser la fraction des dépenses à la charge de 1,3 million de ménages aux revenus modestes.

très incitatif sur le développement du secteur des services à la personne et sur le recours de ces services par nos concitoyens qui en ont le plus besoin.

intitulé et dans la proposition de loi du même jour. Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, et a été porté par des députés issus de plusieurs sensibilités politiques à l'Assemblée cadre du PLF pour 2018. Si l'économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d'échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l'inadaptation de nos règles fiscales et sociales. Celles-ci prévoient, en matière d'impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception, si ce n'est pour les ventes d'occasion et pour le « partage de frais », au champ très restrictif. S'agissant de l'affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales, tout repose sur la distinction entre les particuliers et les professionnels, laquelle n'est, à ce jour, définie par aucun critère simple et objectif. Dans le monde « physique », ces règles étaient en fait largement ignorées pour les petits échanges entre les particuliers, dans le cadre de vide-greniers ou d'autres services occasionnels entre voisins. Mais dans le monde « numérique », où les échanges de pair à pair sont devenus un phénomène massif, et bien souvent traçable et standardisé, ces règles ne sont plus tenables. Si elles étaient appliquées à la lettre, des millions de particuliers de bonne foi seraient pénalisés : mais, comme elles ne le sont pas, de nombreux « faux particuliers » échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels. Il est d'autant plus urgent d'agir que la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne sera obligatoire à partir du 1 janvier 2019. Cet amendement prévoit donc d'instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l'économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 euros. En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 euros par an des plateformes en ligne, soit 250 euros par mois ou 60 euros par semaine, seraient exonérées d'impôt sur ces revenus. Au-delà, l'avantage fiscal serait dégressif et s'annulerait progressivement. Par conséquent, les personnes ayant une activité significative sur Internet seraient imposées sur l'ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence. En matière sociale, le seuil de 3 000 euros 3 000 euros donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un particulier d'un professionnel. Concrètement, l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en deçà de ce seuil plancher, mais elle demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme des professionnels et souhaitent bénéficier d'une couverture sociale à ce titre. L'avantage fiscal serait accordé aux seuls revenus faisant l'objet d'une déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi serait créé un cercle vertueux, permettant d'assurer la juste imposition des activités économiques significatives. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d'impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes

L'amendement que nous proposons est une mesure de clarification et de simplification au bénéfice de tous, réclamée par tous. Il a été excellemment défendu par notre collègue Antoine Lefèvre, s'inspirait d'un rapport que nous avions commis sur la fiscalité de l'économie collaborative, et qui pointait un besoin de simplicité, d'unité et d'équité. Le Gouvernement s'est dit opposé à cette mesure, au motif qu'elle serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt, car elle serait réservée aux utilisateurs des plateformes. C'est une analyse qui nous paraît, pour notre part, contestable, et cette discussion est l'occasion de vous demander des réponses à plusieurs questions précises, monsieur le secrétaire

un avantage fiscal lié à une fiabilisation des déclarations. Ensuite, le principe d'égalité s'apprécie toujours au regard d'autres principes constitutionnels, notamment le principe d'intelligibilité de la loi et le principe de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'ailleurs, le code général des impôts regorge de régimes dérogatoires.

qui a conduit le Sénat, peut-être avant tout le monde, à s'intéresser à la question de l'économie collaborative et aux évolutions de consommation que nous connaissions avec le développement d'Internet. Ce travail a débouché sur un premier amendement,

ces revenus ne sont pas déclarés. J'ai bien entendu notre collègue Julien Bargeton, mais ne se pose pas simplement la question des loueurs d'appartements à Paris, avec Airbnb. C'est toute l'économie collaborative qui se développe, dans tous les secteurs

révolution fiscale importante sur l'économie numérique et l'économie de plateforme, et elle mérite une étude, notamment sur les questions du coût,

avec les opérateurs et les acteurs de cette économie de plateforme, que nous recevons régulièrement, notamment les acteurs liés à l'activité de location meublée et,

qui ne nous paraissent pas toujours justifiées et soulèvent quelques interrogations du point de vue du droit. Il octroie un avantage fiscal au seul motif qu'un revenu est déclaré une plateforme en ligne. De plus, le seuil d'exonération de 3 000 euros va bien au-delà

euros de revenus. Or la Ville de Paris, par exemple, exige que les propriétaires puissent acheter un autre bien s'ils mettent le leur en location- cela figure sur le site de la Ville de Paris.

effet, ce n'est pas la première fois que je présente cet amendement. Il s'agit du problème de la déductibilité des charges supportées par les non-résidents qui tirent de leurs revenus en France l'essentiel de leurs ressources.

Si vous avez le malheur de traverser le détroit de Gibraltar et de vous installer au Maroc ou en Tunisie, vous ne pouvez pas les défalquer.

du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, votre proposition irait au-delà de la jurisprudence administrative récente qui ne concerne que la Suisse du fait des accords passés entre ce pays et l'Union européenne. L'accord sur la libre circulation des personnes, conclu en 1999 entre la Suisse et l'Union européenne, prévoit de tenir compte

des salariés d'une entreprise quand elle soutient la fondation de cette même entreprise. Autant pour les salariés, cela peut se comprendre parce qu'on incite, dans un esprit d'entreprise, les salariés à participer à l'activité d'une fondation qui est celle de l'entreprise. Mais pour les actionnaires, les mandataires sociaux, le sujet est un peu différent, puisque

En même temps, autant le dispositif était justifié pour inciter les salariés, autant, pour les actionnaires qui ont un lien direct avec la politique de la fondation elle-même, cela me paraît un peu plus compliqué.

Dès lors qu'il s'applique aux dons réalisés en 2017 par les mandataires sociaux, les sociétaires, les actionnaires, les adhérents de l'entreprise fondatrice ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, il ne revêt aucun caractère incitatif. Il pourrait

en plus de votre autoconsommation, vous êtes assujettis à la TVA à un taux de 20 %. En revanche, si vous ne faites qu'autoconsommer, vous êtes assujettis à un taux de TVA de 10 %.

3 à 6 kilowatts crêtes afin que nous soyons en situation de favoriser le développement des énergies renouvelables, bien indispensable pour réussir les enjeux de l'accord de Paris.

en dessous duquel les exploitations d'installations photovoltaïques sont soumises à un taux réduit de TVA de 10 % et non au taux normal de 20 %. Pour ce faire, l'amendement se réfère à un seuil

La doctrine administrative admet toutefois qu'un particulier dont la puissance de l'installation photovoltaïque n'excède pas 3 kilowatts crêtes soit présumé comme produisant une électricité intégralement autoconsommée et ne soit pas assujetti à la TVA, ce qui lui permet de bénéficier du taux réduit de 10 % sur son installation photovoltaïque. Contrairement à ce que laissent penser

Personne ne regrettera la taxe d'habitation- en tout cas, pas moi ! Nous en connaissions, évidemment, les limites et l'incapacité pendant des années à la réformer.

clés de cette réforme. Évidemment, ce doit être une invitation à réfléchir à la suite ; nous devons inventer la fiscalité locale moderne de demain. D'ailleurs, le Président de la République l'a dit devant le congrès des maires de France. On parlait à l'instant du numérique. Or la façon dont il bouleverse notre économie et nos villes est aussi, peut-être, une nouvelle ressource à explorer. Il faut, à partir de cette réforme, et au-delà de 2020, bâtir une fiscalité locale moderne, c'est-à-dire

n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. La parole

plus la proportion d'exonérés s'élève dans la population d'une commune, plus nous en savons sur la modestie des ressources des familles. Jusque-là, il n'y

Que l'on ne nous raconte donc pas de bobards ! L'essentiel des catégories populaires de ce pays et les classes moyennes n'auront pas d'amélioration de leur pouvoir d'achat. collègue ! Cela pose la question d'une refonte plus globale de l'impôt local ; je me réjouis que le Président de la République l'ait annoncée.

Deuxièmement, cette promesse de campagne entraîne, contrairement à ce qui vient d'être dit, une amélioration évidente du pouvoir d'achat des Français.

À titre personnel, je suis favorable à la mise en oeuvre de la suppression de la taxe d'habitation de la façon proposée par le Gouvernement. En effet, cela allégera les charges qui pèsent sur les familles les plus modestes, et ce à plus forte raison dans un contexte de hausse de la CSG. l'application de cette mesure pose à l'évidence deux problèmes, qui ont déjà été évoqués. En premier lieu, on ne peut pas imaginer maintenir durablement la taxe d'habitation pour encore 20 % des ménages si l'on s'accorde tous à dire que c'est un impôt injuste.

En somme, la mise en application de cette mesure amorce une réflexion et, sans doute, une réforme plus globale de la fiscalité locale. Le Président de la République l'a d'ailleurs annoncé hier

qu'il ne faut pas s'inquiéter, puisque le Président de la République propose une refonte en profondeur de la fiscalité locale ! C'est donc qu'il revient sur sa promesse de campagne ! J'avoue avoir du mal à comprendre cette langue du nouveau monde, qui consiste à dire en même temps tout et son contraire. C'est la raison pour laquelle, pour

revanche que, sous la V République, le Parlement était chargé d'appliquer strictement les engagements de campagne du Président de la République. Je pensais que la séparation entre le législatif et l'exécutif donnait au Parlement un pouvoir de débat et de vote, même si, là où il y a une majorité en faveur du Président, j'imagine qu'elle vote pour ses réformes. Oui

par construction, mais aussi parce que la révolution fiscale locale mérite d'être amplement engagée. Eh oui ! Elle a déjà commencé. Le gouvernement précédent l'a fait, si j'ose dire, avec le point de TVA que nous avons mis en place dans le projet de loi de finances pour les régions.

termes, vous nous demandez de répondre à votre interrogation institutionnelle, qui n'est pas à sous-estimer et pour laquelle nous pouvons avancer très vite, en nous demandant de ne pas baisser les impôts de nos concitoyens l'année prochaine.

Monsieur le ministre, j'avoue que j'approuve le dispositif, même si j'émets quelques réserves sur ce que vous venez de dire. Si je comprends bien,

qu'un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités sera discuté dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. Cela signifie qu'il n'est pas garanti

toujours mises en oeuvre dans le mois ou les quelques mois qui suivent une élection. Il faut prendre du temps. Je l'ai dit, le Président de la République a une légitimité démocratique incontestable, mais les élus locaux, les maires notamment, qui sont les élus préférés des Français,

Le scrutin est ouvert.

Pour les résidents vivant dans des EHPAD privés non lucratifs non assujettis aujourd'hui à la taxe d'habitation, cette position favorable devrait être pérennisée. À défaut

augmente singulièrement le reste à charge de tous les résidents des EHPAD privés non lucratifs. Par ailleurs, il provoque un ressaut tarifaire dans les quelques EHPAD privés

de statut public. Il s'agit ici de mettre en évidence la différence de traitement entre ces EHPAD qui partagent pourtant les mêmes valeurs de désintéressement et assument les mêmes missions d'intérêt général. Ce rapport permettra certainement d'éclairer cette distorsion et peut-être d'y mettre un terme, si cela est avéré.

de ski implantées sur les bois et les forêts de l'État sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l'utilisation ou de l'occupation du domaine public, par des actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation. Afin d'éviter que ces redevances ne soient fixées de manière trop prohibitive ou hétérogène, le présent amendement vise à encadrer par la loi leurs modalités de mise en oeuvre, de sorte qu'elles ne puissent dépasser un pourcentage préfixé du chiffre d'affaires de la station de ski. Il est prévu que ce pourcentage soit déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme, ce qui permettrait de concilier deux objectifs ne paraissant pas antinomiques : la mobilisation de ressources suffisantes par l'État, ou ses opérateurs, pour la préservation des bois et des forêts, d'une part,

prendre mon cas personnel, j'ai reçu très récemment une offre comprenant un service de presse, assortie d'un prix global.

a sans doute nécessité de réduire les dépenses publiques dans d'autres domaines et de procéder à certaines augmentations de droits indirects, notamment du taux normal et des taux réduits de la TVA. La TVA, qui représente aujourd'hui plus de 50 % des recettes fiscales de l'État, figure largement à la première position s'agissant de nos recettes

Les mêmes qui subissent depuis des années le poids des mesures d'allégement du coût du travail en étant confinés à des niveaux de rémunération faibles sont donc appelés à solder les conséquences de ces choix fiscaux antérieurs. Nous vous proposons, avec cet amendement, de donner un signe pour aller vers une forme de rééquilibrage de notre fiscalité, avec la baisse du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, pour procéder, en compensation, au relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés. Quel

du code général des impôts exonère de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, une minorité de librairies appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises et bénéficiant du label « Librairie indépendante de référence

La situation s'est aggravée par la concurrence de plus en plus vive de la grande distribution ainsi que par la vente de livres en ligne proposée par des plateformes mondiales, qui bénéficient par ailleurs d'un régime fiscal beaucoup plus favorable.

La réforme envisagée ne porte atteinte ni à la liberté des collectivités locales d'appliquer ou non le régime d'exonération prévu par l'article 1464 I du code général des impôts, ni aux finances des collectivités locales concernées, l'accroissement du nombre de librairies qui peuvent, par ailleurs, bénéficier du régime d'exonération étant limité. Quel

Ces amendements tendent à relever le taux de TVA à 10 %, contre 5,5 % actuellement, pour l'acquisition de terrains à bâtir, la construction et la rénovation d'immeubles dans le secteur du logement social.

4,2 millions de logements HLM, occupés par plus de 10 millions de personnes, et 15 % des ménages, dont la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté, relèvent du logement social. Pratiquant un loyer moyen de 390 euros, contre 570 euros dans le parc privé, les organismes d'HLM répondent déjà à une forte demande sociale.

Nous espérons vraiment que le Gouvernement et le Président de la République nous entendront. La parole est à M. le ministre.

souhaitons attirer l'attention sur la nécessité de trouver des moyens d'aider le financement de logements intermédiaires, tant dans les quartiers prioritaires de la

Le régime des BRS a été créé voilà un an dans une optique de lisibilité et de stabilité de la norme fiscale. N'ayant pas le recul nécessaire sur sa mise en oeuvre, je ne crois pas opportun de changer la norme fiscale.

de 10 %, pourvu que les titulaires de ces droits démembrés respectent les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour que l'immeuble lui-même bénéficie du taux intermédiaire. L'amendement est donc partiellement déjà satisfait : je ne peux que confirmer les propos de mon prédécesseur.

au taux réduit de TVA de 10 %, tout programme de construction de logements intermédiaires doit comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes

pourraient proposer des loyers inférieurs de 20 % aux loyers de référence sur le marché libre et développeraient un dispositif d'usufruit locatif institutionnel s'appuyant sur les offres de vente des pavillons des particuliers concernés.

Cet amendement a pour objet d'atténuer les distorsions de concurrence qui existent entre le secteur de l'hôtellerie, soumis à la TVA, et celui de la location de meublés touristiques, qui en est exonéré. De fait, la France a une interprétation très restrictive de la notion de fonction similaire à celle de l'hôtellerie, prévue notamment par la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. En France, pour être assujetties à la TVA, les locations de meublés touristiques doivent en effet être accompagnées d'au moins trois prestations proposées par les hôtels : service de petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge Cette transposition du droit européen antérieure à l'explosion de la location de logements par l'économie collaborative n'est à l'évidence plus adaptée à la réalité du secteur. Échappent ainsi à la taxation les personnes qui mettent à disposition des meublés touristiques, la plupart du temps pour des locations de courte durée. Ainsi, pour rétablir une égale et saine concurrence entre les hôtels et les locations de meublés touristiques, on pourrait introduire, comme l'a fait l'Allemagne par exemple, un critère unique qui serait fonction de la durée de la location. Ce critère serait d'ailleurs plus conforme au droit de l'Union européenne, la Cour de Justice de l'Union européenne l'ayant elle-même jugé plus pertinent.

à la journée, à la semaine ou au mois sont supérieurs à 23 000 euros seront affiliés au régime social des indépendants, ce qui réduira la concurrence malsaine que vous évoquez, madame la sénatrice. Ces particuliers sont donc désormais redevables des cotisations sociales, comme tout hôtelier.

ou la prestation d'un service en direction de l'un ou l'autre des États ou territoires dits « non coopératifs » sur le plan fiscal, les ETNC, c'est-à-dire, en langage moins technocratique, les « paradis fiscaux ». Nous préférerions que